Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

alors que près de 10 milliards d'êtres humains pourraient peupler le monde d'ici à trente ans, les systèmes alimentaires qui se sont développés dans les pays occidentaux au XX siècle, et largement diffusés depuis sur la planète, sont aujourd'hui problématiques. Ils posent en effet des questions en termes de santé, de consommation de ressources naturelles, d'impacts sur le climat et de préservation de la biodiversité. Ils sont d'ailleurs de plus en plus contestés, soulevant des oppositions croissantes sur les plans éthique, social et politique, mais aussi quant à leur soutenabilité et à leur efficacité économique réelle. De manière accrue aujourd'hui, la problématique de l'indépendance protéique de la France et de l'Europe devient centrale, alors que la crise du covid-19 a mis en exergue les effets désastreux pour les populations que pourrait provoquer la rupture des circuits mondiaux d'approvisionnement. Nous avons pu constater pendant le confinement, notamment dans nos départements, le succès des circuits court, agriculture paysanne (AMAP), le désir de manger sain et, plus globalement, l'importance de définir des plans territoriaux en matière d'alimentation. Le rôle de premier plan des collectivités locales est ainsi souligné. Il est donc aujourd'hui nécessaire de rechercher quelles inflexions et quelles ruptures pourraient permettre de faire émerger des systèmes alimentaires plus durables. Cela a été l'objet du long travail que j'ai mené avec mon collègue sénateur du Finistère, Jean-Luc Fichet, pendant près de six mois, donnant lieu, le 28 mai dernier, à la présentation d'un rapport contenant vingt propositions.

Premièrement, nous voulons remettre la sécurité d'approvisionnement alimentaire au coeur des politiques publiques et assurer un meilleur équilibre des apports animaux et végétaux, notamment par le développement des légumineuses, visant ainsi une autonomie protéique. souhaitons associer plus étroitement éducation, santé et environnement, à travers des déclinaisons nationales d'un programme européen Nutrition santé et environnement. Il s'agit de prévenir, d'une part, les maladies de pléthore, c'est-à-dire manger trop et mal, et les risques de dénutrition, pas manger assez, et, d'autre part, s'adapter au réchauffement climatique en préservant la biodiversité. Je rappelle à ce propos que l'alimentation, du champ à l'assiette, représente près de 25 % de l'empreinte carbone des ménages français. Troisièmement, il s'agit de lutter contre les inégalités sociales d'accès à une alimentation de qualité, en actionnant les leviers financiers, à travers les aides et les fonds européens, les leviers éducatifs, et ceux de la formation et de la recherche. voulons encourager le développement de la filière des légumineuses, qui semble être la clé de voûte du type de transition alimentaire souhaitable et souhaitée aujourd'hui, plus sobre et plus végétale. Le 20 mai 2020, la Commission européenne a présenté aux institutions européennes sa stratégie « De la ferme à la fourchette ». Les recommandations clés de ce plan portent cette ambition forte de bâtir une « chaîne alimentaire bénéfique pour les producteurs, les consommateurs, l'environnement et le climat », dans le cadre du Pacte vert européen, et en lien avec la défense de la biodiversité. Le rapport partage au final la plupart

je me félicite de la tenue de ce débat sur les conclusions de notre rapport, qui a reçu un écho important et des retours très positifs à la suite de sa publication, le 28 mai dernier. principales propositions pour aller vers une alimentation plus durable est de renforcer la lutte contre les inégalités sociales face à l'alimentation. Les études montrent que c'est surtout dans les milieux modestes que l'on retrouve les régimes ayant le plus d'effets négatifs sur la santé et l'environnement. Il existe donc aujourd'hui un véritable clivage social en la matière : le taux d'obésité parmi les ménages les plus modestes est ainsi plus de quatre fois supérieur à celui qui est observé Outre les causes économiques de ces inégalités, sur lesquelles je vais revenir, il nous faut également tirer les leçons du bilan mitigé des politiques de recommandations nutritionnelles menées depuis vingt ans. Il est temps de passer à une véritable éducation au mieux manger, qui associe un dépistage et un suivi nutritionnels renforcés, afin d'accompagner les ménages pour mieux choisir, mieux acheter, mieux préparer. Compte tenu du coût des pathologies liées à une alimentation non saine, cette éducation à l'alimentation durable sera un investissement plus que profitable pour la collectivité. Il est en outre indispensable d'accompagner l'éducation et la responsabilisation individuelle des consommateurs par un réel effort d'assainissement de leur environnement alimentaire. On ne peut pas à la fois financer des campagnes d'information et tolérer que les aliments les plus aisément accessibles soient les plus déséquilibrés sur le plan nutritionnel. Nous attendons de véritables engagements de tous les professionnels de l'alimentation, et il faut avoir le courage de défendre certaines mesures concrètes. Nous devons par exemple aller sans ambages vers la reformulation des recettes des plats industriels. Certaines entreprises ou marques ont déjà pris ce virage. Mais les aliments transformés restent dans l'ensemble beaucoup trop gras, beaucoup trop sucrés et beaucoup trop salés. Ils regorgent aussi trop souvent d'additifs dont les effets de long terme sur la santé sont source d'inquiétudes. Soyons clairs : il ne s'agit pas de diaboliser l'industrie agroalimentaire. Compte tenu de nos modes de vie, les aliments transformés industriellement garderont une place centrale. Mais c'est une raison de plus pour assainir cette offre sur le plan nutritionnel Nous préconisons par ailleurs de rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel et environnemental des aliments. C'est un dossier de niveau européen, et la France doit se mobiliser à ce sujet ! Le Nutriscore est en effet un outil puissant pour aider les consommateurs à identifier les aliments les plus sains et inciter les producteurs à assainir leur offre. offre. Le combat contre une alimentation qui nuit à la santé et à l'environnement ne peut pas négliger la question des prix. Les aliments qui composent un régime sain sont en effet généralement les plus onéreux. Les fruits et les légumes frais coûtent plus cher que le sucre et la graisse. Le poisson frais n'est pas accessible à de nombreuses bourses. pour les aliments bio. Comment espérer que nos concitoyens les plus modestes leur donneront plus de place alors qu'ils sont déjà ceux qui consacrent à l'alimentation l'effort budgétaire le plus important ? Lutter contre les inégalités face à l'alimentation durable est une question de justice, mais aussi de pragmatisme. Pousser les consommateurs à manger durable, c'est en effet inciter agriculteurs, industriels et distributeurs à transformer leur offre. La transition alimentaire du XXI siècle, qui est la clé d'une population et d'un environnement en meilleure santé, sera tirée par la demande.

En 2020, tout récemment, hier matin, la Convention citoyenne pour le climat, dont le Président de la République a reçu les membres, a mis au coeur de sa réflexion trois : alimentation, environnement et transition agroécologique.

Mais, soyons honnêtes, avant cette crise dramatique du covid-19, que nous avons traversée et que nous traversons encore, nul ne pouvait imaginer que l'alimentation

Nos enseignes de distribution, qu'il est facile de critiquer, ont été à la hauteur. Elles se sont adaptées et ont permis à leurs clients, c'est-à-dire à nos concitoyens, d'acheter les denrées alimentaires qu'ils souhaitaient.

devons encore travailler sur ce sujet. Enfin, vous évoquez évidemment la malnutrition et la précarité économique et sociale. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une alimentation à deux vitesses dans notre pays,

Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

l'un des leviers pour concrétiser l'objectif d'alimentation durable tracé dans les lignes de ce rapport consiste sans doute à valoriser l'agriculture française et son excellence, notamment la proximité, lorsque cela est possible. La crise que nous venons de traverser ne fait que conforter cette affirmation. Les secteurs agricole et alimentaire sont à la croisée de plusieurs domaines dont l'importance est grandissante. Je veux bien sûr parler d'une alimentation saine et de qualité pour tous nos concitoyens, d'un niveau de vie décent pour nos agriculteurs, mais aussi, entre autres, de l'impact du changement climatique, de la modernisation des méthodes grâce au numérique ou encore des progrès techniques et technologiques. Cela me

certes nécessaire de respecter les grands principes de la commande publique, mais il faut aussi simplifier les règles d'accès aux marchés publics

Le modèle d'agriculture à la française, par ses multiples visages qui ont été évoqués- petites fermes, grandes fermes, intensif et extensif -, est celui de l'équilibre le plus soutenable et le plus résilient. l'a dit en classant, trois années durant, le modèle d'agriculture français comme le plus durable.

parmi les plus bas, et qui se débattent toujours contre une concurrence déloyale imposée par les accords de libre-échange, notamment l'accord économique et commercial global (CETA). Pouvez-vous donc nous expliquer, monsieur le ministre, en quoi le CETA est compatible avec nos objectifs de souveraineté, de résilience alimentaire et de neutralité carbone ? Partout en France, nos agriculteurs cultivent la terre. C'est la singularité de notre pays. Pourtant, il existe des territoires où la terre est moins fertile. Quelle PAC demain pour ces agriculteurs des zones dites intermédiaires, ceux qui s'épuisent à cultiver et à entretenir des zones à faible rendement, contribuant ainsi à une agriculture de proximité

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise nous a rappelé que, pour relever le défi de l'alimentation durable, nous devions renforcer notre résilience alimentaire. Or, depuis 2000, vous le savez, notre alimentation sous toutes ses formes dépend de plus en plus d'importations. C'est le cas par exemple de la viande de volaille, importée pour

Faire venir du poulet de l'autre bout de l'Europe, nourri avec des protéines qui contiennent des OGM américains ou brésiliens, alors que la France était un producteur majeur voilà quelques années : on marche sur la tête ! Contre cette politique, oui, il faut relocaliser nos productions, mais il faut pour cela être en capacité de rendre notre alimentation accessible à tous les consommateurs, quel que soit leur pouvoir d'achat. Or, si la France a aujourd'hui un modèle agricole qui permet de garantir des denrées alimentaires de grande qualité, accessibles à tous, c'est parce que la PAC, dès sa constitution, a souhaité soutenir les agriculteurs pour leur permettre d'être compétitifs, parfois en vendant au-dessous des coûts réels de production,

c'est prendre le risque de ne réserver les produits français, à forte valeur ajoutée, qu'à certains, condamnant les plus modestes aux produits importés, moins chers, mais sans aucune garantie de cohérence avec nos normes de production. C'est aussi priver nos producteurs de la plus grosse partie du marché. L'alimentation durable ne peut pas s'opposer à une alimentation accessible à tous. Ma question est donc simple, monsieur le ministre : que compte faire le Gouvernement pour la compétitivité de notre agriculture sur les produits d'entrée de gamme ?

la crise économique et sociale due à la crise sanitaire nous oblige à repenser nos modes de production et de consommation. Les enjeux sont nombreux et tous primordiaux, au nombre desquels s'impose le devoir de tendre vers un système plus vertueux, plus soucieux de l'environnement, de la biodiversité et de la qualité des sols. Au cours d'enquêtes, nos concitoyens expriment clairement ces préoccupations et revendiquent l'accès à une alimentation de qualité, durable et locale. Les nombreuses auditions que j'ai coanimées sur ce thème au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable démontrent, de façon évidente, qu'il faut repenser notre modèle agricole. La crise pandémique a révélé la fragilité de la chaîne alimentaire et notre dépendance à certains produits, posant la question non seulement de la sécurité alimentaire, mais aussi de la souveraineté. Répondre à ces deux priorités, sécurité et souveraineté, c'est poser aussi la question du bien manger. Cela suppose de reconsidérer les pratiques agricoles, mais aussi de bâtir une vraie politique alimentaire à l'échelle des territoires. Il est indispensable d'accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique et numérique. Il est indispensable aussi de relocaliser l'agriculture, de soutenir les producteurs locaux et de développer une polyculture urbaine. Il faut aider à l'installation de jeunes agriculteurs, alors qu'un agriculteur sur deux va partir à la retraite dans les dix ans. Mais cela ne peut s'envisager qu'au moyen d'une politique foncière volontariste, permettant l'accès à la terre. Cela justifie la grande loi sur le foncier que le Président de la République lui-même avait appelée de ses voeux au salon de l'agriculture en 2019. Vous venez, monsieur le ministre, de l'évoquer et d'en confirmer la nécessité.

La concurrence de l'agriculture française n'est pas internationale ; elle est à 95 % ou 98 % européenne. Tant que nous ne réglerons pas

Cette opinion, partagée sur les travées du RDSE, se concrétise notamment dans le travail effectué par notre collègue Françoise Laborde dans sa proposition de résolution sur la résilience alimentaire, déposée en décembre dernier. Dans ses travaux, elle souligne le caractère indispensable à la vie de la Nation du foncier agricole, mais aussi la nécessité de renforcer la capacité d'anticipation et de prévention des pénuries. Elle fait également le lien entre résilience alimentaire et sécurité nationale, en proposant une révision de la loi de programmation militaire pour réfléchir à l'intégration de la production alimentaire et du foncier agricole nourricier comme secteur d'activité d'importance vitale. Pour revenir à des considérations plus locales, le problème qui se pose aux territoires ruraux, c'est une double mécanique qui voit, d'une part, la réduction des terres agricoles et, de l'autre, la hausse du prix du foncier, deux vrais freins à l'installation de nouvelles exploitations, et donc à la construction de notre souveraineté alimentaire. Qu'on le veuille ou non, la crise que nous venons de vivre nous a rappelé que cette idée de souveraineté alimentaire française, voire européenne, était assez difficile à intégrer, avec un nombre conséquent de produits que nous importons. Oui, monsieur le ministre, il faudra continuer le travail de pédagogie sur la nécessité de manger local et de saison, mais cela sera vain sans une véritable impulsion donnée par l'État. Récemment, et je m'en réjouis, le Président de la République a fait sien le terme de souveraineté alimentaire. Aussi, monsieur le ministre, comment comptez-vous adapter la PAC pour vous donner les moyens de vos ambitions ?

le plus urgent, aujourd'hui, c'est un plan de relance pour éviter qu'il y ait des centaines de milliers de chômeurs d'ici à la fin de l'année. C'est la priorité du Gouvernement. Sur le foncier, le Président de la République s'est exprimé hier- il suffit de l'écouter -, rappelant

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons nous rappelle toute l'importance de la sécurité alimentaire et du besoin de savoir que l'on pourra s'alimenter en qualité et quantité

un véritable statut et d'en faire définitivement un secteur d'activité d'importance vitale. Sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, garantie d'un accès à une alimentation de qualité pour nos pour nos concitoyens, notamment les plus précaires, préservation de la biodiversité, voilà les piliers qui doivent inspirer des contrats alimentaires territoriaux passés avec les collectivités.

véritables bassins de vie, à un horizon raisonnable, 2022. Ils doivent aussi faire l'objet de révisions régulières. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas faire des EPCI des autorités organisatrices de l'alimentation durable et locale ? Le contrat territorial doit affirmer le primat de l'alimentation durable et de notre sécurité alimentaire comme outil de développement de développement par tous et pour tous. Les collectivités territoriales en ont la volonté et elles ont montré ces dernières semaines à quel point elles étaient essentielles pour la vie quotidienne de nos concitoyens. N'attendons pas 2050 pour repenser notre alimentation ! C'est ce à quoi nous ont invités les cent cinquante membres de la Convention citoyenne ont fait de l'alimentation durable et locale l'un des axes de leurs propositions. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que le contrat alimentaire territorial doit être, demain, un outil essentiel pour cultiver ensemble notre jardin et faire vivre notre exception alimentaire aujourd'hui plus qu'essentielle ?

qui passe par une relance de la production de la luzerne pour la nourriture animale. Une telle nourriture permet de produire de la viande et du lait riches en carotène et en oméga 3, ce qui est bon pour la santé des Français.

Les protéagineux sont naturellement riches en protéines, alors que nous achetons du soja transgénique en masse en provenance d'Asie et d'Amérique du Sud. Favoriser leur développement permettrait d'avoir des produits plus sains et éviterait de les importer de l'autre bout du monde, ce qui réduirait l'empreinte carbone. De plus, ils s'intègrent facilement dans la cuisine traditionnelle française qui fait notre renommée internationale. Une alimentation durable ne passe pas uniquement par du bio, mais avant tout par une alimentation diversifiée, équilibrée et de proximité.

La résilience de notre modèle agricole et agroalimentaire pendant la crise sanitaire du coronavirus devrait nous pousser à remercier et à respecter nos agriculteurs,

On pourrait croire que le seul but est de détruire l'agriculture française ! Pour cela, nous ne sommes pas à une contradiction près. Quand vous proposez de végétaliser l'assiette des Français, en demandant de manger moins de viande et donc plus de fruits et légumes, et quand dans le même temps vous souhaitez que la France retrouve plus d'autonomie alimentaire, vous ignorez- plutôt, encore plus grave, vous faites semblant d'ignorer -que nous sommes autosuffisants en viande, alors que nous importons un fruit et un légume sur deux,

Elle nous interroge aussi sur nos proximités de solidarité, nos modes de production et de consommation et leurs impacts environnementaux. L'approche territoriale semble évidente pour partager une stratégie, définir en commun les objectifs et s'en donner les moyens.

outre, en matière d'aménagement foncier et de politique d'urbanisme, la singularité alimentaire est négligée et le manque de spécifications est à noter. Au même titre que les plans ne serait-il pas souhaitable de généraliser la mise en oeuvre de plans d'alimentation durable au sein des EPCI qui pourraient ainsi les déléguer, par intégration territoriale, dans les PAT ? Dans ce cas, un axe logistique est forcément nécessaire afin d'organiser les circuits locaux et compléter les approvisionnements de proximité pour livrer les donneurs d'ordre dans les meilleures conditions.

Ces propositions s'appuient sur l'existant et contribuent à renforcer la territorialité. L'appropriation de ce sujet et son acceptabilité par les acteurs seraient acquises- le département de la Gironde est par exemple prêt à accompagner les collectivités sur ces questions. Qu'envisagez-vous concrètement sur ces sujets ?

il y a près de soixante ans, ici même au Sénat, le ministre de l'agriculture, Edgard Pisani, présentait la loi d'orientation agricole qui porte son nom et qui faisait suite à d'autres dispositifs importants adoptés deux ans plus tôt. Élaborée en lien avec Michel Debatisse, leader des jeunes agriculteurs, cette loi devait répondre aux faiblesses relevées à l'époque : « bas niveau de vie, absence d'espoir, vie difficile pour les femmes, inaptitude à la vie économique moderne ».

avec, entre autres, des démarches de qualité- IGP, AOP, AOC, agriculture biologique, label rouge, etc. -qui rassurent les consommateurs et sont le fer de lance de notre industrie agroalimentaire, si puissante à l'export. Monsieur le ministre, le Président de la République a parlé hier de souveraineté alimentaire. Par conséquent, envisagez-vous de proposer une nouvelle loi d'orientation agricole qui permette aux agriculteurs et éleveurs de réellement vivre de leur métier et en même temps d'assurer à nos concitoyens une alimentation de qualité la plus locale possible

Pour aller vers une alimentation durable, ce rapport nous invite, en premier lieu, à répondre à l'enjeu de l'autonomie alimentaire que notre pays a perdue au fil des dernières décennies. La crise due au covid-19 a permis de mesurer notre état de dépendance à l'égard d'acteurs d'acteurs lointains dans de nombreux secteurs stratégiques, particulièrement en matière d'alimentation. Cette indépendance est une question vitale, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour notre planète. Elle doit être un objectif de court terme pour préparer dès aujourd'hui les grands défis qui s'imposent à nous à l'horizon de 2050 : atteindre la neutralité carbone et nourrir une population de 10 milliards d'êtres humains

notre collègue Françoise Laborde a soutenu une proposition de résolution sur la résilience alimentaire des territoires qui soulevait la question de l'autonomie alimentaire. Elle pointait du doigt la grande dépendance de nos territoires qui ne maîtrisent qu'une partie infime des ressources agricoles consommées directement par leur population : 2 % en moyenne dans les cent premières aires urbaines. Pourtant, ces aires urbaines disposent localement des moyens pour couvrir plus de 54 % des besoins de la consommation alimentaire de leurs habitants. Si l'autarcie alimentaire complète des territoires n'est pas réalisable ni même souhaitable, l'objectif d'un degré d'autonomie de 50 % est tout à fait atteignable. Il ne manque aujourd'hui que la volonté politique pour organiser la reconnexion entre production et consommation de produits agricoles. Le rapport préconise ainsi de soutenir et d'encourager les projets alimentaires et agricoles de territoire afin d'accroître la part des approvisionnements locaux dans la consommation régulière.

faut définir le modèle agricole agroalimentaire que l'on veut pour notre pays, mais cela ne peut pas se faire uniquement à l'intérieur de la France. Notre pays est un timbre-poste à l'échelle de la planète.

Mme Catherine Dumas. Je veux tout d'abord remercier et féliciter nos collègues Cartron et Fichet pour la qualité de leur rapport. Pour ma part, j'aimerais profiter de ce débat en faveur d'une alimentation durable pour attirer votre attention, monsieur le ministre, sur le grave problème de dénutrition, qui est devenu un véritable enjeu de santé publique dans notre pays. On parle de dénutrition lorsque les apports alimentaires sont insuffisants pour couvrir les besoins nutritionnels des personnes. En France, on estime à 2 millions le nombre de cas. J'étais hier en réunion de travail avec des chefs, comme Christian Têtedoie, Michel Guérard, mais aussi des parlementaires, engagés comme moi sur les dossiers liés à la table française, des médecins nutritionnistes ou exerçant auprès des personnes âgées ou de grands malades. Il ressort de nos discussions que ce que l'on peut baptiser « malbouffe » à l'hôpital touche 10 % des enfants malades, 20 % des adultes hospitalisés, et ce chiffre grimpe à 40 % chez les patients cancéreux, et plus de 50 % chez les personnes âgées hospitalisées. (Ehpad), un tiers des résidents auraient besoin de mieux se nourrir. La dénutrition a des conséquences concrètes mesurables. On constate une augmentation de la durée de séjour à l'hôpital, des réadmissions non programmées et de la mortalité. La dénutrition à l'hôpital, c'est d'abord un problème de budget on dispose rarement de plus 4 euros de coût matière pour préparer le petit-déjeuner, le déjeuner, un goûter et le dîner. C'est aussi un problème de formation : les personnels qui travaillent en restauration collective ne sont pas toujours sensibilisés aux problématiques.

sénatrice. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le rapport d'information de nos collègues dresse un état des lieux du système alimentaire français et formule des propositions pour faire émerger une alimentation plus durable. L'une de ces propositions consiste à promouvoir un discours équilibré et apaisé sur la consommation de produits animaux : il faut en manger moins pour manger des produits de meilleure qualité. C'est une volonté qui fait son chemin chez bon nombre de nos concitoyens. Comme vous le savez, l'élevage extensif répond parfaitement à ce double objectif du moins et du plus. En montagne, par exemple, les animaux élevés en plein air rejoignent les alpages aux beaux jours pour redescendre dès les premières gelées. gelées. Ils entretiennent l'espace, contribuent à la biodiversité et les produits qui en sont issus, la viande, le lait et le fromage, ont un intérêt nutritionnel incontestable.

En effet, les bergers sont contraints de parquer leurs troupeaux, de les rentrer le plus souvent possible dans les bergeries, et de réduire, d'année en année, la période d'estive. Alors, forcément, la qualité de la viande s'en ressent. C'est bien dommage C'est bien dommage pour les amateurs de l'agneau de Sisteron, par exemple, car il pourrait bientôt disparaître de nos boucheries. L'Union internationale pour la conservation de la nature précisait, en 2014, dans son rapport sur les écosystèmes montagnards montagnards : « La labellisation implique des normes de qualité et de fabrication qui imposent de conserver les procédés traditionnels d'élevage et les méthodes artisanales de production à la ferme. Elle favorise ainsi souvent les pratiques de parcours qui permettent de maintenir ou de créer des paysages agricoles ouverts, favorables à la biodiversité. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si l'élevage extensif a encore un avenir en France. Quelles sont les perspectives d'avenir crédibles pour ces éleveurs,

En 2050, il y aura 10 milliards d'humains sur terre. Les besoins alimentaires vont donc être multipliés par deux. Face à cette réalité, notre pays doit être responsable, innovant et exemplaire.

4 milliards de repas chaque année. Ce sont donc des acteurs clés du secteur. Depuis la loi Égalim, l'idée d'une gouvernance territoriale partagée par l'ensemble des acteurs du système agricole et alimentaire reste un concept assez mal défini,

ne doit pas être discriminante en fonction de la situation économique, sociale ou géographique. Elle doit être la même pour tous, et c'est ce que je nous engage à viser collectivement. Réfléchissons à une souveraineté alimentaire européenne, qui passe d'abord par une souveraineté alimentaire française,

pour une meilleure alimentation : manger sain et durable, et que nos producteurs locaux puissent trouver à s'épanouir. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce débat.